La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Il n'y a pas

L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote du projet de loi de finances pour 2020, adopté par l'Assemblée nationale (projet Avant de passer au vote sur l'ensemble du texte, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits par les groupes pour expliquer leur vote. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents,

La justice fiscale est renforcée au travers de la baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu au profit des classes moyennes, qui se traduira par un gain moyen de pouvoir d'achat de près de 300 euros pour 17 millions de foyers fiscaux.

La démarche de « sincérisation » du budget se poursuit, l'amélioration de la lisibilité du système fiscal progresse, avec le toilettage de nombreuses niches et microtaxes. Nous nous en réjouissons. ce budget pour 2020 a donné le coup d'envoi de la réforme de la fiscalité locale, selon des modalités finalement assez proches de celles qu'avait pu formuler notre commission des finances. Je pense en particulier à la revalorisation des valeurs locatives dans le cadre du droit en vigueur. Je pense aussi au renforcement du mécanisme de garantie du montant des fractions de TVA affectées aux départements. En tout cas, la réforme paraît bien calibrée pour ne pas répéter les erreurs du passé. Avec des fortunes diverses, le groupe Union Centriste a contribué au débat sur la réforme de la fiscalité. L'occasion nous est donnée ici de saluer la mise en place du simulateur LexImpact, dont nous espérons la pérennisation et l'extension, à l'avenir, à d'autres impôts que l'impôt sur le revenu.

J'en viens à la seconde partie du projet de loi de finances. Le groupe Union Centriste a soutenu l'adoption de la grande majorité des missions budgétaires. La stabilisation ou la légère baisse des crédits consacrés à la plupart d'entre elles constitue un effort louable dans un contexte délicat pour nos finances publiques.

à but éducatif, culturel et sportif. Quant aux articles non rattachés, ils ont fourni l'occasion de débats

ayant un lien avec le développement durable et l'écologie le même jour constitue un progrès, il n'est pas possible à mon sens de travailler sur ce sujet lors de l'examen d'un projet de loi de finances ni même lors de celui de la loi sur l'économie circulaire. circulaire. Nous devrions programmer un débat spécifique sur la fiscalité verte pour avoir davantage de lisibilité et de compréhension, tant les dispositifs sont variés et multiples et les interventions des uns et des autres diverses et parfois contradictoires. Sur l'initiative conjointe de notre commission des finances et de la commission du développement durable, nous pourrions organiser un tel débat, qui serait certainement extrêmement productif.,

que le dispositif antifraude aux dividendes, que nous avions déjà adopté l'année dernière et que l'Assemblée nationale avait complètement vidé de sa substance, sera cette fois-ci maintenu en l'état. Ce serait une victoire de l'optimisme sur l'expérience

monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, mes premiers mots seront pour remercier notre rapporteur général et les services de la commission des finances. Chacun mesure la charge de travail qu'a représentée l'exercice avec près de 2 500 amendements examinés Le Sénat va donc se prononcer sur le budget tel qu'il a été modifié lors de nos débats. Monsieur le secrétaire d'État, je ne saurais trop vous conseiller, comme l'année dernière et la précédente, si ce n'est sur tous les sujets- ne rêvons pas ! -, au moins sur certains, de tenir compte des votes du Sénat. Je commencerai bien sûr par nos collectivités territoriales en rappelant d'ailleurs qu'elles demeurent le seul bon élève de la classe en matière de contribution au redressement des finances publiques.

et maintenant un gel, c'est-à-dire un effort supplémentaire, d'environ 10 % sur le quinquennat, inflation comprise. Ce n'est pas rien ! Alors, au moins, donnons-leur de la visibilité. Vous supprimez la taxe d'habitation et coupez ainsi le lien démocratique que représente la contribution au financement des services publics locaux pour une bonne moitié des habitants de nos communes. Nous avons fait le choix d'amender votre texte pour nous donner le temps d'en mesurer les conséquences, notamment en ce qui concerne les dotations de péréquation. Rien ne serait pire en effet que de revivre un épisode tel que celui que nous avons connu avec la refonte de la carte intercommunale.

Nous avons également sécurisé la fraction de TVA que percevront les départements. Nous avons rendu aux communes le produit des exonérations de taxe sur le foncier bâti accordées par la loi aux bailleurs sociaux, mais payées en fait par les communes.

Pour les familles, grandes oubliées de votre politique, nous avons approuvé la baisse de l'impôt sur le revenu, mais nous avons, comme chaque année, souhaité faire un geste significatif en faveur du quotient familial pour 1,4 million de foyers fiscaux. Nous avons porté à 70 000 euros le plafond de l'abattement fiscal des donations aux petits-enfants, afin d'encourager la solidarité intergénérationnelle. pour la transition énergétique (CITE) aux propriétaires bailleurs, accordé des avantages fiscaux pour le verdissement des flottes automobiles des entreprises et prévu des mesures de suramortissement pour certains équipements.

: nous ne pouvons plus alourdir les impôts de production, fût-ce pour financer des projets importants. Du côté des dépenses, pour vous aider à trouver des économies, sujet sur lequel vous êtes à la peine, nous avons augmenté le temps de travail dans la fonction publique en l'alignant sur la moyenne du privé,

En seconde partie, les débats nous ont conduits à repousser les crédits de missions importantes telles que la justice, la sécurité, l'immigration, l'agriculture et l'écologie.

ce projet de loi de finances pour 2020 tel que le Sénat l'a modifié, mais sans se faire beaucoup d'illusions sur ce que fera l'Assemblée nationale. En fait, ce texte marquera bien l'acte II du quinquennat, celui du renoncement au retour à l'équilibre de nos comptes publics. En 2018, comme en 2017, la France était toujours championne des prélèvements obligatoires dans l'OCDE avec un taux inchangé de 46 %. En 2019 et en 2020, une baisse devrait s'amorcer, mais au prix d'un déficit du budget de l'État supérieur à 90 milliards d'euros, alors qu'il s'élevait à 67 milliards d'euros en 2017 et à 76 milliards d'euros en 2018, sans parler des comptes de la sécurité sociale qui vont replonger dans le rouge. nous découvrirons peut-être le prodige par lequel le Premier ministre mettra en oeuvre une réforme des retraites qui devrait, selon ses mots, ne faire aucun perdant, mais beaucoup de gagnants, sans reculer l'âge de départ et sans creuser davantage le déficit, pourtant déjà annoncé entre 10 et 17 milliards d'euros en 2025, c'est-à-dire demain. Gageons malheureusement que le train de l'État continuera de rouler vers l'abîme de la dette. Mes chers collègues, notre cher et vieux pays est certes difficile à réformer mais, pour avoir une chance d'y parvenir, il faudrait de la pédagogie, de la méthode et le courage de dire la vérité aux Français. Pour ce qui est de la pédagogie et de la méthode, les dernières semaines laissent penser que l'agence du père Ubu a pris le contrôle de la communication du Gouvernement. Quant au courage, craignant qu'il vous ait manifestement abandonné, je terminerai en citant Clemenceau : « Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire ; quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, autant le dire tout de suite : ce projet de loi de finances confirme l'abandon par ce gouvernement de tout objectif de redressement à moyen terme de nos comptes publics.

vous faites pourtant bien pire, alors que vous avez bénéficié d'une croissance bien meilleure. Tout en abandonnant l'objectif de redressement

qui touchent plus de 1 200 euros de retraite, ou encore non-indexation des retraites sur l'inflation. Alors, c'est vrai après avoir essayé de capter 9,5 milliards d'euros de recettes, et pour ne pas avoir écouté le Sénat qui vous avait pourtant clairement mis en garde sur les conséquences possibles de telles mesures, dû reculer en désordre, soit pour renoncer à ces recettes, soit pour financer en catastrophe une batterie de mesures pour un coût total évalué à ce jour à 17 milliards d'euros. On en voit le magnifique résultat, qui doit tout à votre savoir-faire politique.

Malgré de meilleures recettes fiscales, malgré de moindres dépenses grâce au taux d'intérêt de la dette, vous gagez ce remboursement en ne prenant pas en charge le coût des mesures « gilets jaunes » dans le budget de la sécurité sociale, pour un coût estimé à 3,5 milliards d'euros. Pour imager un peu votre politique, vous bouchez les trous en en recréant d'autres à côté. J'ai eu récemment l'occasion de dire que cela me faisait furieusement penser aux Shadoks,

mais simplement en les faisant financer par la dette ou en recréant artificiellement un déficit de la sécurité sociale, ne saurait ramener la confiance. Il en est de même de l'ensemble des réformes que vous avez mises en oeuvre à marche forcée et qui affaiblissent le pouvoir d'achat des Français, souvent les plus fragiles 700 millions d'euros d'économies sur la seule année 2020 pour l'assurance chômage, 1 milliard d'euros sur les APL notamment. Ne vous étonnez donc pas, monsieur le secrétaire d'État, si vous ne bénéficiez plus aujourd'hui de la compréhension populaire suffisante pour entreprendre de nouvelles réformes. Je l'ai dit : sur la taxe carbone, sur la non-indexation des retraites et sur la CSG, le Sénat vous a mis en garde. L'écouterez-vous davantage aujourd'hui qu'en 2019 ?

Cette réforme présente encore trop d'angles morts auxquels il est possible de répondre si l'on s'en donne le temps. Des amendements corrigeant les problèmes les plus simples ont été votés ici.

Compte tenu de leur importance, un an de travail supplémentaire ne sera vraiment pas de trop. Je me réjouis par ailleurs que le Sénat ait réindexé plusieurs prestations sociales sur l'inflation. Nous espérons que ces amendements seront repris définitivement par le Gouvernement. Effectivement, on peut toujours espérer, comme le disait notre collègue Dallier. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce budget pour 2020 se distingue par l'abandon de toute volonté de redressement des comptes publics, par de nombreux rétropédalages traduisant une méconnaissance profonde des aspirations de nos concitoyens par une incapacité à construire l'avenir conjointement avec le Parlement. Monsieur le secrétaire d'État, le ministre de l'économie nous avait dit ici, en 2017, qu'il avait une boussole ce gouvernement a donc une boussole. Il ne lui manque donc plus qu'à définir un cap ! Vous l'aurez compris, notre groupe votera contre ce projet de loi de finances.

l'examen du projet de loi de finances marque chaque année un moment intense de la vie parlementaire. Il est même historiquement au coeur de notre légitimité de représentants de la Nation. L'actualité s'y invite aussi, venant parfois perturber le déroulement très strict et contraint de la discussion. L'histoire a tout de même tendance à se répéter. L'an dernier, alors que notre pays était secoué par la crise des « gilets jaunes », le Président de la République annonçait les mesures d'urgence économiques et sociales destinées à y répondre la veille du vote solennel du Sénat sur le budget. Aujourd'hui, nous nous réunissons à nouveau pour ce vote solennel, alors que le Gouvernement s'apprête demain à faire des annonces importantes concernant le projet de réforme des retraites. J'observe également que l'examen de la première partie a été complexe,

L'éligibilité des propriétaires bailleurs au CITE va dans le sens d'une incitation plus forte à la rénovation énergétique des logements, alors que ce secteur demeure en France celui qui a le plus de progrès à effectuer en matière de modernisation, de transition écologique et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Je me félicite par ailleurs de l'adoption d'amendements présentés par les membres de mon groupe, comme celui relatif à la taxe sur les surfaces commerciales des, celui concernant la sécurisation des petites lignes aériennes, chère à Josiane Costes, ou encore ceux sur l'énergie et les carburants. Le Sénat a également entériné l'abaissement à 11 % de la deuxième tranche de l'impôt sur le revenu. Cette baisse devrait en réalité s'accompagner de recettes supplémentaires grâce au prélèvement à la source. L'impôt sur le revenu et la fiscalité du patrimoine suscitent toujours d'importants débats. Le groupe du RDSE est traditionnellement attaché à l'idée d'impôt citoyen qu'incarnait à l'origine l'impôt sur le revenu,

Le lien entre impôt et citoyenneté s'est malheureusement abîmé, ce que nous déplorons. Peut-être faut-il y voir la raison de la crise du consentement à l'impôt sur laquelle je m'étais déjà exprimé l'an passé. Dans le domaine de la fiscalité des entreprises, si les gros acteurs tirent leur épingle du jeu, les petits rencontrent plus de difficultés, en particulier du fait de la diversité des régimes applicables. On peut ainsi regretter que n'aient pas été adoptés certains amendements tendant à harmoniser les régimes d'imposition des bénéfices pour les micro-entreprises, en particulier les micro-exploitations agricoles. La seconde partie n'a pas compté moins d'amendements ! L'année dernière constituait déjà un record. C'est le revers de la normalisation du collectif budgétaire de fin d'année le PLF est désormais le seul texte de l'automne où l'on puisse déposer des amendements fiscaux, ce qui est fidèle à l'esprit, mais conduit à une certaine inflation du nombre d'amendements. Mais nous sommes là dans notre rôle de législateurs de plein exercice Eh oui ! S'agissant des aspects les plus positifs, je note, pour ma part, le doublement des crédits alloués à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, dont la création est due à une initiative de notre groupe, ainsi que la revalorisation à 10 millions d'euros de la prime d'aménagement du territoire. Sur d'autres missions, nous avons également rencontré quelque succès, comme la revalorisation de 2 points de la retraite des anciens combattants, défendue par Nathalie Delattre, ou encore le déplafonnement de la dotation aux bourgs-centres, défendu par Maryse Carrère. La défense des intérêts des départements est également un axe de notre politique, avec la préservation de leurs ressources propres, comme les produits des droits de mutation, en particulier dans les départements ruraux, mais aussi dans la grande couronne de la région parisienne. Je salue enfin la prorogation du prêt à taux zéro en zone rurale, dans les conditions fixées par l'article 50 , dont la possible suppression avait suscité de nombreuses inquiétudes. Toutefois, ces éléments ne peuvent faire oublier le rejet d'autres propositions, comme l'élargissement de l'assiette de l'impôt sur le revenu, la TVA réduite sur des produits de première nécessité, ou encore une nouvelle répartition du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau. Plus largement, comment se prononcer sur un budget amputé de cinq missions- et non des moindres, puisque sont concernés la justice, l'intérieur ou encore l'agriculture ? Les raisons du rejet de ces crédits sont parfois légitimes, parfois plus simplement partisanes

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission, que je tiens à mon tour à remercier, mes chers collègues,

une série de débats techniques, intéressants et, souvent, pertinents, mais force est de constater que, à l'issue de ces débats, les grands équilibres du texte n'ont pas été modifiés. L'article 2 relatif à la baisse d'impôt sur le revenu n'a pas été supprimé. L'article 5 portant réforme de la taxe d'habitation a été maintenu. L'article 11 tendant à réduire l'impôt sur les sociétés n'a pas été rejeté. L'article 16 visant à supprimer le taux réduit de TICPE sur le gazole non routier a été voté. La refonte des taxes sur les véhicules à moteur de l'article 18

impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, fiscalité écologique, lutte contre la fraude fiscale, aucune grande orientation de ce texte n'a été

se fait le porte-voix des corps intermédiaires, qu'il appelle à leur respect, vous allez d'un trait de plume, sans même engager une négociation avec les organisations syndicales, remettre en cause les conditions de travail et la rémunération des agents.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les conséquences dévastatrices de l'entêtement du Gouvernement semblent ne pas vraiment lui sauter aux yeux ! Un avertissement électoral sévère en mai, des grèves et un mouvement des « gilets jaunes » qui persistent, des manifestations de pompiers, d'avocats, de paysans et de policiers, dont le nombre de suicides est toujours plus important. Une insécurité qui grandit, des Français qui travaillent, mais qui n'arrivent plus à boucler leurs fins de mois ou à survivre avec leur maigre allocation de retraite. Mais rien de toute cette misère, de toute cette France de la souffrance ne vous fait changer d'avis, monsieur le secrétaire d'État. Enfermé dans votre bunker de Bercy, vous imposez l'austérité, à la recherche du moindre sou qui resterait au fond de la dernière poche des travailleurs, des familles et des retraités. L'Élysée, de son côté, refuse de recevoir notre collègue rapporteur de la mission « Pouvoirs publics » pour le Sénat ... C'est un scandale ! Un rapport sur les agapes d'un Emmanuel Macron et de ses apôtres ne serait sans doute pas le bienvenu en ces temps d'hyper-austérité, quand on sait, déjà,

Votre trajectoire budgétaire est désastreuse. Dans le même temps où vous exigez des Français qu'ils se serrent la ceinture- quand elle a encore des trous pour ce faire ! -, vous prévoyez d'accroître les dépenses des ministères de 6,6 milliards d'euros. C'est de l'auto-engraissement étatique, au détriment du muscle économique dont nos compatriotes ont pourtant Par ailleurs, les belles promesses printanières Par ces engagements venus des ministères Et qui étaient autant de bourgeons exemplaires Laissent la place à un automne lapidaire Où les fruits pourris des promesses non tenues Accablent les Français aujourd'hui dans la rue. Sur le plan de la justice, une loi printanière promettait des crédits en augmentation. Il manque aujourd'hui 150 millions d'euros à la trajectoire votée. Sur le plan de la sécurité, nous ne voyons aucune augmentation de crédits qui aurait permis la création de nombreux postes dont nous avons besoin pour reconquérir ces fameux territoires perdus de la France, de la France française ! Sur le plan migratoire, c'est toujours le même paradigme : les autres avant les nôtres ! Cumulant ce qui se fait de pire à droite, avec la déréglementation tous azimuts, dans une concurrence mondiale, donc déloyale, avec ce qui se fait de pire à gauche, avec l'hyper-fiscalité qui ruine les ménages et plombe nos entreprises, triste et surtout inquiétante est l'image d'un corps étatique impuissant, impotent et même schizophrène Mais, cette année encore, Noël ne vous offrira pas le miracle que vous attendez ... Vous souhaitiez une France « en marche », monsieur le secrétaire d'État ; elle l'est ! Elle marche dans les rues de France et de Navarre pour vous faire savoir qu'elle en a assez de votre politique, de votre stratégie, qui consiste à facturer, à fracturer, à mépriser, à diviser. Je voterai, par conséquent, contre ce projet de loi de finances, qui n'est que la énième traduction de la position d'un gouvernement refusant toute alternative à sa ligne d'austérité généralisée.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, quel singulier télescopage entre ce jour de vote du projet de loi de finances au Sénat et les innombrables rassemblements et manifestations qui se déroulent, en ce moment même, dans notre pays pour la défense de notre système de retraites par répartition Ces journées de mobilisations font suite à l'année ininterrompue de manifestations au cours desquelles nos concitoyens réclamaient plus de justice sociale, plus de justice fiscale. En un mot : les moyens de mener une vie décente dans cette société. d'État, vous l'avez souvent méprisé et vous avez beaucoup manoeuvré pour tenter de contenir cette colère légitime. Il est temps de changer votre logiciel. Durant ces dizaines d'heures de débat, la phrase que nous avons entendue le plus est la suivante : « Il faut réduire la dépense publique. formule a été répétée à l'envi par les uns et les autres dans cet hémicycle. Certes, ce gouvernement a su faire assaut de communication pour vendre à l'opinion que ce budget était celui du pouvoir d'achat rendu à nos concitoyens. L'année 2018 restera l'année durant laquelle 400 000 de nos concitoyens auront basculé dans la pauvreté. L'Insee indiquait dans son rapport annuel que le taux de pauvreté atteignait désormais 14,7 % de la population française. Quel incroyable paradoxe de compter dans ce pays, sixième puissance économique mondiale, 9 millions de gens vivant sous le seuil de pauvreté À vrai dire, la stratégie de communication du Gouvernement, axée sur la hausse du pouvoir d'achat et la protection de l'environnement, ne trompe personne. L'écart entre vos discours et la réalité n'a jamais été aussi prononcé Même vos alliés centristes du Modem à l'Assemblée nationale s'inquiètent, dans une tribune récente, de l'aggravation de la situation. Je vais me permettre de les citer Il y a consensus sur les origines du mal : dans une mondialisation désordonnée et surtout dérégulée, le capitalisme provoque plus que jamais des inégalités grandissantes. grandissantes. Chaque Français sent bien que la croissance générale profite principalement à quelques-uns. » Et plus loin : « Force [ ...] est de constater que, durant l'année des gilets jaunes, les distributions de dividendes ont battu leur record historique et que les émoluments des patrons du CAC 40 ont crû de 14 %. Qu'on soit de droite, du centre ou de gauche, cette seule énonciation provoque l'indignation, explique la révolte. » Franchement, mes chers collègues, nous n'avons rien à modifier à ce propos ; un éditorial du quotidien n'aurait pu mieux dire vous demandez toujours plus d'efforts à nos administrations, aux collectivités et aux Français, mais, dans le même temps, vous confirmez les cadeaux aux plus fortunés. Pendant le quinquennat, vous aurez procédé à plus de 197 milliards d'euros d'allégements fiscaux en faveur des plus aisés et des grands groupes. Le constat tiré de ce projet de loi de finances est, lui, sans appel : pratiquement toutes les missions budgétaires sont victimes de coups de rabot. L'un des grands perdants n'est autre que Bercy. Les annonces de suppressions de postes n'ont cessé de pleuvoir, à tel point qu'entre 2020 et 2022 pas moins de 5 775 d'entre eux auront disparu. Pendant ce quinquennat, 10 500 postes de fonctionnaires d'État, tous départements confondus, auront été supprimés. C'est sans précédent ! Franchement, au moment où la Cour des comptes rend un rapport cinglant sur l'efficacité de votre lutte contre l'évasion fiscale, vous feriez bien d'y réfléchir à deux fois Les débats au Sénat n'auront pas permis de modifier la nature profonde de ce budget. Ce n'est pas le sympathique amendement de notre rapporteur général visant à créer l'impôt sur la fortune improductive, nouvelle mouture de l'IFI, ... Une bonne idée ! ... qui instillera, dans notre système fiscal, un peu plus de la justice fiscale tant attendue par nos concitoyens. Notre groupe avait proposé en première partie le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), la suppression de la à l'heure où les dividendes s'envolent, la mise en place d'un barème de l'impôt à 11 tranches avec un taux maximal de 65 %. Toutes ces mesures concrètes ont été balayées sans sourciller. Les transferts de crédits décidés ici ou là, à enveloppes fermées, n'apporteront pas non plus de mieux-être à nos concitoyens. Quelques millions en plus pour les maisons de l'emploi ou ceux accordés aux collectivités pour la restauration du patrimoine ne pourront apporter plus d'efficacité aux missions budgétaires.

D'ailleurs, nous avons noté que la majorité sénatoriale, jamais en reste sur de nombreux sujets fondamentaux, profite de ce projet de loi de finances pour faire voter une série d'amendements très rudes pour les fonctionnaires, en imposant, par exemple, trois jours de carence et en allongeant au passage le temps de travail. Nul doute que les agents de la fonction publique hospitalière sauront apprécier à sa juste mesure le message fort que cette majorité souhaite leur envoyer ... Au fond, les différences entre le Gouvernement et la majorité sénatoriale sont de l'ordre de la nuance.

Cette proposition aurait dû faire l'objet d'un rejet global, tant elle est un mauvais coup supplémentaire porté à l'autonomie financière des collectivités et au principe de libre administration ! Nous aurions ainsi pleinement joué notre rôle d'assemblée des collectivités territoriales.

Voici la première : « Le capitalisme du XX siècle n'est plus viable. La croissance ne peut plus se faire au prix d'une destruction de la planète et de l'explosion des inégalités au sein d'un même pays. »

...] dans la commune que réside la force des peuples libres. » Tocqueville ! « Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la mettent à la portée du peuple ; elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Sans institutions communales, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de la liberté. » d'Alexis de Tocqueville n'ont rien perdu de leur pertinence. Ils trouvent dans cet hémicycle, au sein de la chambre des territoires, un écho plus puissant qu'ailleurs. si le Sénat s'attache à défendre les institutions communales, et leur autonomie financière, c'est d'abord par la conviction qu'elles se trouvent au fondement de notre démocratie. Alors que nous nous apprêtons à nous prononcer sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2020, cette conviction nous oblige tout particulièrement. Elle nous oblige parce que ce budget, qui doit lancer l'acte II du quinquennat, redéfinit assez largement les contours de la fiscalité locale. Sous l'allégorie de la prudence, qui veille sur les travées de notre assemblée, nous devons faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande exigence. Prudence, vigilance, exigence : je crois que ces trois mots ont guidé notre action tout au long de l'examen de ce budget et, singulièrement, lorsqu'il s'est agi de veiller à l'autonomie financière et à l'attractivité économique de nos territoires. Sur certains sujets, mes chers collègues, nous avons su afficher une opposition constructive, et ce pratiquement à l'unanimité du Sénat. C'est notamment le cas pour la rationalisation du mécénat d'entreprise : l'approche comptable proposée par l'article 50 n'a pas convaincu sur ces travées. Nous savons ici que le mécénat permet bien souvent de faire émerger, au niveau local, des synergies entre collectivités territoriales, entreprises et associations. Comme cela a été rappelé lors du débat organisé par notre groupe, ici même, en mai dernier, le mécénat de proximité s'avère trop précieux à nombre de nos territoires pour que le Sénat se risque à en rationaliser le dispositif. Cette rationalisation rimerait avec complexification et désaffection. La simplicité constitue, en l'occurrence, un gage d'efficacité ! Il ne faut pas se tromper de combat : on ne réduira pas notre déficit public en rabotant à la marge des dispositifs qui structurent l'économie de nos territoires. Nous avons su en apporter la preuve en défendant certaines politiques qui participent à la cohésion de nos territoires, sans dégrader l'équilibre budgétaire du projet de loi initial. Ainsi, l'amendement que j'ai défendu avec ma collègue Sophie Taillé-Polian au nom de la commission des finances, visant à augmenter de 5 millions d'euros les crédits alloués aux maisons de l'emploi, va dans le sens d'un maillage plus solidaire de nos politiques en faveur de l'emploi. Sur d'autres sujets, nous nous sommes montrés plus conciliants, en amendant les articles votés à l'Assemblée nationale. C'est notamment le cas pour l'article 51, qui instaure une taxe forfaitaire sur les CDD d'usage. Nous sommes nombreux sur ces travées à avoir rappelé qu'on ne lutte pas contre la précarité en taxant davantage l'emploi. La solution que nous soutenions, et qui a été retenue par la commission, visant à repousser d'un an l'entrée en vigueur de cette taxe paraît ainsi raisonnable. Nous espérons qu'elle sera conservée dans la loi de finances et qu'elle permettra une négociation Mais ce n'est pas toujours faire preuve de sagesse que de repousser d'un an la mise en oeuvre des réformes. Je pense ici à l'article 5 ... En modifiant en profondeur le financement des collectivités locales, il a fait l'objet de longs débats et cristallisé les oppositions politiques. Nous avons su y apporter des améliorations très importantes, comme la revalorisation des valeurs locatives au niveau de l'inflation. Mais, au final, une majorité d'entre nous cherchent à gagner du temps dans l'application de cette réforme. Or il ne s'agit plus de nous prononcer sur le principe de la suppression de la taxe d'habitation. Cette décision a été validée par les urnes. Elle est attendue par nos concitoyens. Je crois, pour ma part, qu'il ne faut plus en retarder la mise en oeuvre. J'entends que ce report se fera sans incidence pour le contribuable et qu'il s'agit simplement de garantir le financement des collectivités territoriales. Bien évidemment, mon groupe partage cet objectif. Cependant, c'est aussi ignorer les chantiers qui sont devant nous en matière de fiscalité locale, notamment pour ce qui concerne les impôts de production. En effet, même si ce projet de loi de finances allège globalement la pression fiscale sur les ménages et sur les entreprises, le chemin qui reste à parcourir est encore long. Nous accusons encore, notamment vis-à-vis de notre voisin allemand, un manque de compétitivité flagrant, et les impôts de production pèsent lourdement dans la balance. Je pense ici à la contribution économique territoriale, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, au versement transport. Tous ces impôts se trouvent aujourd'hui au fondement de l'autonomie financière des collectivités territoriales, mais ils grèvent notre économie. Pour donner suite à l'engagement pris par le Président de la République de réduire cette pression fiscale qui freine l'investissement dans les territoires, pour répondre aux attentes des entrepreneurs qui s'obstinent à vouloir produire en France, en Anjou, dans les Mauges, et ce sans diminuer les ressources des collectivités territoriales, le Sénat doit proposer plus que temporiser. Il faut même accélérer sur certains sujets, notamment pour réduire le déficit public et résorber notre dette. En ces temps de relative accalmie, il est clair que nous n'allons pas aussi vite que nous le devrions, compte tenu du retard que nous avons accumulé pendant des décennies. Certes, l'objectif d'un déficit contenu sous la barre des 3 % semble désormais acquis, et on a tôt fait d'oublier les efforts consentis pour cela. Mais il faut maintenant redoubler d'ambition et viser le déficit zéro Cette ambition ne se fonde pas sur une vision morose d'un État rabougri. Bien au contraire ! Il s'agit de trouver les voies et moyens de renforcer l'État dans ses fonctions régaliennes, de le doter d'une armée, de forces de l'ordre et d'une justice à la hauteur des défis de ce siècle. Mais cette ambition, sous la contrainte de la rigueur budgétaire, suppose que nous puissions collectivement redoubler d'efforts dans les prochaines années. Pour conclure, mes chers collègues, ce budget, tel que l'a amendé le Sénat, poursuit la baisse des prélèvements obligatoires, tout en respectant l'autonomie financière des collectivités locales et la maîtrise du déficit public. Je crois qu'il va donc dans la bonne direction. Mais nous le privons d'ambition en cherchant à gagner du temps. Nous l'avons aussi privé d'ambition, monsieur le président,

le scrutin public est de droit. Conformément à l'article 60 du règlement, il va être procédé à un scrutin public à la tribune,

Elle n'est qu'en partie liée à la croissance du nombre d'articles à examiner, puisque le texte transmis par nos collègues de l'Assemblée nationale n'a- si je puis m'exprimer ainsi -augmenté que de 50 % en deux ans. En tout état de cause, nous ne disposons toujours que de vingt jours pour examiner l'ensemble du PLF, avec, de surcroît, l'examen au sein de cette période du projet de loi de

sachant que nous constatons aussi une augmentation sensible du nombre d'amendements sur les missions budgétaires et les articles qui leur sont rattachés, augmentation supérieure à 50 % en deux ans. À l'avenir, il nous faudra tenir ces délais, tout en veillant à ne pas dégrader les conditions de notre examen parlementaire. Enfin, en cet instant, je voudrais surtout remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce travail collectif : l'ensemble des membres du Gouvernement et M. le secrétaire d'État, qui se sont succédé en séance et à la tribune, et leurs collaborateurs, avec lesquels nous avons plaisir à travailler vous-même, monsieur le président du Sénat, ainsi que les vice-présidents de notre assemblée, qui ont été très sollicités. Je salue particulièrement M. le rapporteur général, qui a été le plus mobilisé d'entre nous en cette période, ici même dans l'hémicycle, sur la banquette maintes fois évoquée,

le service de la séance et celui de la commission des finances, ainsi que nos collaborateurs politiques et les professionnels de nos groupes, qui ont été particulièrement actifs. Merci à chacun d'entre vous.

d'achever cette première lecture de la loi de finances. Je voudrais particulièrement remercier mes collègues qui, sur toutes les travées, ont fait preuve de compréhension

pour les relations à la fois constructives et courtoises que nous avons pu entretenir, et que nous entretenons de manière générale tout au long des débats. Certains désaccords ont pu être exprimés entre la majorité du Sénat et le Gouvernement, parfois entre le Sénat- vous l'avez dit -et le Gouvernement. Je forme le voeu que, malgré ces désaccords, nous puissions, sur un certain nombre de points, continuer à avancer. Deuxièmement, vous me permettrez de mettre à profit- si j'ose dire -le fait que le Gouvernement ne participe pas à la commission mixte paritaire, pour dire que je ne préjuge pas de son résultat, et que je ne peux ni le prévoir ni le commander.